à M. le secrétaire d'État. Il s'agit d'actualiser les montants des compensations au titre des transferts de compétence des régions et des départements, et donc de modifier les fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ou TICPE, pour un ajustement total de 7,7 milliards d'euros.

Monsieur le rapporteur général,

emploi », « Administration générale et territoriale de l'État » et « Justice » au titre des transferts prévus aux collectivités territoriales. Il s'agit du transfert de la gestion des fonds européens aux régions ; du transfert de la compensation aux régions des dépenses de personnel transférées en application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,

chargés de la gestion du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, transférés au 1 janvier 2015 ; enfin, du transfert au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnel transférées dans le cadre de la décentralisation des Centres de L'amendement technique n° 231 modifie, lui, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Il procède à plusieurs corrections des compensions versées aux départements et aux régions, en particulier les régions d'outre-mer, afin de traiter les compétences pour lesquelles les compensations sont portées sur le programme « Concours financiers aux collectivités territoriales car elles ne peuvent faire l'objet d'une compensation par la voie de l'affectation de TICPE. Il majore donc la dotation générale de décentralisation affectée aux départements au titre des corrections des compensations prévues dans le cadre des transferts de services du ministère de la transition écologique et solidaire liés à la loi de 1985. Il majore également la dotation générale de décentralisation affectée aux régions au titre, d'une part, des corrections des compensations prévues dans le cadre de la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes introduite par l'arrêté du 2 septembre 2015 et, d'autre part, de la compensation prévue au titre des services chargés des compétences transférées aux régions par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Il majore enfin les concours particuliers de la dotation générale de décentralisation au titre des corrections des compensations prévues dans le cadre du transfert des services du ministère de la transition écologique et solidaire, chargés de la gestion des ports départementaux et des ports d'intérêt national, de la gestion des aérodromes, en application de la loi LRL, ainsi que de la gestion du domaine public fluvial

Il est très largement concentré sur les salaires du secteur privé, les traitements de la fonction publique, les pensions versées par l'État et les retraites de la sécurité sociale.

Enfin, la prévention de la fraude fiscale, qui pourrait animer la réforme, n'est pour nous guère justifiée, puisque l'impôt sur le revenu est loin d'être le plus fraudé. En 2016, sur les 15 292 millions d'euros de droits simples rappelés après contrôle fiscal, 4 028 millions 4 028 millions concernaient l'impôt sur les sociétés, 2 433 millions les taxes sur le chiffre d'affaires et 2 203 millions les droits d'enregistrement et l'impôt de solidarité sur la fortune. On comptait 2 397 millions d'euros de droits rappelés en matière d'impôt sur le revenu, le tout pour 3 350 euros de redressement moyen en matière d'impôt sur le revenu, pour près de 10 000 euros en matière d'impôt sur les sociétés et plus de 8 500 euros en matière de TVA.

le Gouvernement a demandé à l'Inspection générale des finances de mener un audit sur les modalités de mise en oeuvre du prélèvement à la source, son impact sur les contribuables et sur les entreprises. Cet audit, comme le rapport sur les solutions alternatives, confirme que le prélèvement à la source s'avère, à nos yeux, bien plus favorable pour les contribuables que l'actuelle mensualisation ou que les solutions alternatives. En ce qui concerne les entreprises, il confirme que la charge reste limitée, en particulier grâce au déploiement de la déclaration sociale nominative. Le Gouvernement considère que le présent article améliore les conditions de mise en oeuvre de cette réforme en 2019, répond aux recommandations formulées par l'IGF et vise à alléger les modalités et les règles de gestion pour les collecteurs, sécuriser le déploiement de la réforme et conforter l'intérêt des contribuables pour cette réforme. En supprimant cet article, vous pénaliseriez les collecteurs, qui se préparent activement à la mise en place de cette réforme dans les meilleures conditions, et vous supprimeriez les pistes de simplification à leur profit et au profit des contribuables. Le Gouvernement demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, il

dans le cadre de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source. Cette réforme conduit à faire de l'année 2018 une « année blanche », mais cela ne doit pas avoir pour effet de « désinciter » les ménages à réaliser des travaux sur l'année 2018. Pour remédier à cette difficulté, le PLFR soumis au Parlement prévoyait, pour le passage à l'année blanche, d'aligner le traitement des monuments historiques sur celui qui est applicable aux immeubles locatifs de droit commun. Ainsi, les charges de travaux déductibles au titre de l'année 2019 seraient forfaitairement constituées de 50 % des montants respectivement supportés au titre des années 2018 et 2019. Malheureusement, si un tel dispositif a du sens pour les charges de droit commun, sa transposition aux monuments historiques priverait les ménages de toute contrepartie fiscale aux surcoûts précités liés aux travaux supportés en 2018, ce qui les inciterait à ne faire aucune dépense. De surcroît, le mécanisme de pondération pour 2019, conduisant à faire la moyenne avec les dépenses de 2018, réduirait en conséquence de 50 % la prise en compte des dépenses de 2019 : les ménages ne réaliseraient donc pas plus de travaux cette année-là. Il en résulterait donc, pour les monuments historiques, deux années sans travaux : 2018 et 2019. Les conséquences seraient catastrophiques pour la conservation des monuments et pour l'ensemble des entreprises spécialisées de ce secteur du BTP. Pour remédier à cette situation, la commission des finances de l'Assemblée nationale avait adopté un amendement permettant de se rapprocher au plus près de l'objectif, commun au Parlement et au Gouvernement, de réduire autant que possible l'impact de l'instauration du prélèvement à la source, afin de ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux au cours de l'année de transition. En séance publique, devant l'Assemblée nationale, le ministre Gérald Darmanin a fait état de deux difficultés à propos de cet amendement : d'une part, contrairement à son objectif, sa rédaction pouvait avoir des conséquences sur l'ensemble des déficits fonciers de droit commun, et pas seulement sur les dépenses liées aux monuments historiques ; d'autre part, elle pouvait rendre possible une seconde prise en compte des dépenses de 2018 en 2019 et 2020, engendrant ainsi une double déduction injustifiée. Pour ces motifs, l'Assemblée nationale a rejeté

cas bénéficier aux autres immeubles. D'autre part, l'option offerte, permettant de répartir, pour moitié, les dépenses de 2018 sur les années 2019 et 2020, ne permet aucun cumul. Cette solution permet de conserver la prise en compte normale de la réalisation de travaux en 2018 et en 2019, au seul léger inconvénient près, pour les ménages, de reporter pour la première moitié d'un an et pour la seconde de deux ans l'imputation des dépenses réalisées en 2018. La neutralité du passage au prélèvement à la source

du Gouvernement et par voie d'amendement, un dispositif qui permet de préserver totalement les réductions et crédits d'impôt liés aux dons, notamment les dons aux oeuvres, au titre de l'année 2019. Le

d'abord, pour tenir compte des particularités inhérentes à la relation de travail pouvant exister entre le particulier employeur et son salarié, par exemple du fait de l'absence d'un logiciel de paie, des modalités simplifiées de mise en oeuvre de la réforme sont d'ores et déjà prévues. Ainsi, le particulier employeur n'aura aucune relation nouvelle à entretenir avec l'administration fiscale. Il conservera son interlocuteur habituel dans le cas de l'utilisation des kits simplifiés, à savoir pour la garde d'enfants, le Centre national CESU pour les autres emplois à domicile et la mutualité sociale agricole pour les particuliers employeurs employant des salariés agricoles pour une durée de moins de 3 mois et utilisant le titre emploi simplifié agricole. Ce sont ces interlocuteurs qui transmettront l'ensemble des informations déclarées par le particulier employeur- nom du salarié et montant de la rémunération -à l'administration fiscale, en lieu et place de l'employeur. Ces organismes communiqueront au particulier employeur le salaire net de retenue à la source à verser à son employé. L'employeur n'aura donc aucune démarche complexe à effectuer, ni détermination de l'assiette imposable ni calcul de la retenue à opérer sur le salaire. Il ne sera donc exposé à aucun risque d'erreur. Les trois interlocuteurs Pajemploi, centre prélèveront directement sur le compte bancaire du particulier employeur, en plus des cotisations sociales, le montant de la retenue à la source, puis reverseront les sommes ainsi prélevées à l'administration fiscale. En outre, afin de simplifier la vie des particuliers employeurs, ces centres proposeront une option tout-en-un, qui permettra aux employeurs de s'acquitter du paiement du salaire auprès de son salarié par l'intermédiaire des organismes. La proportion des salariés de particuliers employeurs non imposables est estimée à 75 %. L'impact de la retenue à la source pour les particuliers employeurs doit donc être relativisé. Au-delà, l'Agence centrale travaillent actuellement à l'encouragement à la dématérialisation du dispositif CESU en effectuant une campagne de promotion. Afin d'accompagner les employeurs dans leur démarche, est également prévue la mise en place de partenariats avec des relais locaux tels que La Poste ou les maisons de services au public. Pour les particuliers employeurs qui effectuent actuellement leur déclaration sociale par voie papier,

Aujourd'hui, ces primes de jeu sont taxées une première fois au moment de leur perception à un taux de 15 %. Néanmoins, lorsque le joueur se réinscrit l'année suivante au même tournoi, il doit se

Par ailleurs, cette taxation en deux temps induit des charges de personnel importantes. Ainsi, pour le tournoi de Roland-Garros, les organisateurs sont obligés d'installer un bureau fiscal sur place avec trois personnes mobilisées pendant six semaines. De manière à simplifier la législation et à rendre nos événements sportifs internationaux plus attractifs, il est proposé d'instaurer un prélèvement libératoire de 20 % au moment de la perception de la prime. Cet amendement est soutenu par les différentes fédérations sportives concernées. Quel est l'avis de la commission ?

d'euros. Cette somme est soumise à une retenue de 315 000 euros, imputable sur son impôt sur le revenu, lequel serait, pour un célibataire, de l'ordre de 920 000 euros s'il est salarié ou de 1,160 million d'euros s'il est indépendant ou non-adhérent d'un organisme agréé. Avec le système que vous proposez, ce contribuable serait uniquement redevable d'une retenue à la source libératoire de 378 000 euros, ce qui se traduirait, dans l'hypothèse où il est indépendant, par une division de son imposition par trois. Et si le

Autoriser une mobilisation immédiate du crédit d'impôt auprès d'un établissement financier du secteur privé faciliterait l'accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français, dont les foyers les plus modestes, accentuerait la lutte contre le travail non déclaré, entraînerait une simplification des procédures fiscales et permettrait un renforcement de la lutte contre la fraude. Cet amendement s'inscrit dans l'universalisation du crédit d'impôt, puisque la mobilisation immédiate de la trésorerie en résultant concernerait tous les foyers, qu'ils soient imposables ou non. Un organisme consolidateur se chargera de vérifier les informations et de consolider les dépenses mobilisées pour s'assurer du non-dépassement des plafonds de la part des ménages, qui pourront bénéficier de ce dispositif directement ou indirectement, c'est-à-dire dans le cadre de l'emploi direct de personnel ou par le recours à des entreprises ou associations prestataires de services à la personne. Enfin, il convient de souligner que ce dispositif est à coût constant pour l'État, puisqu'il permettra une mobilisation immédiate des crédits d'impôt par les établissements financiers, avec restitution par l'État dans les délais habituels de la liquidation de l'impôt sur le revenu, et donc sans requérir d'effort financier de la part de l'État en termes de montant ou de calendrier de paiement. Quel

liste des actifs bénéficiant d'une exonération partielle de l'impôt sur la fortune immobilière afin de tenir compte de la situation spécifique des propriétaires de monuments historiques. Ceux-ci supportent, en effet, des charges pour l'entretien et la restauration des biens immobiliers dont ils sont propriétaires. En raison de l'intérêt public de conservation, il apparaît nécessaire de prévoir un abattement représentatif des charges et sujétions spécifiques aux monuments historiques, lorsque certaines conditions sont réunies.

l'article 156 du code général des impôts relatif au régime fiscal des monuments historiques ; une affectation de l'immeuble, totale ou partielle, à une activité commerciale ou professionnelle ou à la visite payante, c'est-à-dire en quelque sorte une contribution du monument à l'économie touristique du territoire. Sous ces conditions, il nous paraît normal d'exonérer les propriétaires de l'impôt sur la fortune immobilière.

pour faire en sorte que ce dispositif puisse s'appliquer comme prévu par le texte initial au Nord et au Pas-de-Calais dès le 1 janvier 2018. Le Gouvernement s'est également engagé à continuer de travailler sur la question de la Lorraine.

de tenir une promesse du gouvernement précédent, mais je crains que son honneur ne se limite aux limites de son fief électoral ! Oh ! Je le regrette vivement.

Il prévoit une exonération totale d'impôt sur le revenu pour les traitements et salaires versés par les établissements de santé implantés en ZRR aux médecins y exerçant leur activité pendant cinq années, puis une exonération dégressive sans plafonnement du bénéfice de l'avantage fiscal

Il est destiné à définir un modèle fiscal applicable au projet Cigéo de stockage des déchets nucléaires à haute et moyenne activité et à vie longue.

Une mission IGA-IGF a remis, en mars 2017, un rapport sur le modèle fiscal de Cigéo. Cette mission a estimé que l'utilisation de la taxe de stockage constitue le meilleur levier. Le produit de levier. Le produit de cette taxe spécifique aux installations de stockage de déchets radioactifs peut être réparti de manière flexible entre les collectivités territoriales, sans que les règles de droit commun de répartition de la fiscalité directe

pour accroître le volume de redistribution ; étendre le périmètre de redistribution de la taxe de stockage aux départements et aux régions d'implantation ; enfin, diminuer le de manière analogue à ce qui existe pour d'autres projets à caractère exceptionnel comme le centre spatial de Kourou ou l'usine marémotrice de la Rance, afin de compenser la hausse de la taxe de stockage. Comme cela a été proposé par la mission IGA-IGF,

sans le soumettre aux commissions compétentes, ce qui avait suscité des réactions assez passionnées des uns et des autres. Cependant, cet amendement n'est pas complètement neutre et pose deux problèmes majeurs, ce

Ce dispositif, créé en 2006, fonctionne bien. Il a bénéficié à 110 entreprises en 2016, et il contribue incontestablement à la vitalité de l'industrie française de la musique,

secrétaire d'État. L'article 13, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, étend l'exonération prévue par le I de l'article 1040 du code général des impôts aux acquisitions des établissements publics fonciers de l'État, en complément de l'exonération déjà prévue pour les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance. Le présent amendement apporte deux précisions additionnelles au régime applicable à certains établissements publics d'État : d'une part, l'application de l'exonération aux établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance est clarifiée ; d'autre part, est également clarifié le régime spécifique applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévu par l'article par l'article 1040 Ainsi, en plus de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1040, ces derniers bénéficient d'une exonération de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts. Ces deux précisions permettent d'assurer dans de bonnes conditions le transfert de propriété de l'État aux universités, conformément à loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

Les droits de mutation comprennent les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, et sont dus à l'occasion du changement de propriétaire d'un immeuble, d'un terrain, d'un titre de société ou d'un fonds de commerce. L'amendement vise les mutations d'immeuble. Si le bien est ancien, les droits de mutation payés sont compris entre 5 % et 5,8 % du prix de vente. Ils comprennent la taxe départementale de publicité foncière, les frais d'assiette et de recouvrement au profit de l'État et la taxe additionnelle au profit de la commune. Si le bien est considéré comme neuf, les droits de mutation sont plus faibles, à hauteur de 0,7 %, recouvrant la taxe départementale de publicité foncière et les frais d'assiette et de recouvrement au profit de l'État. La vente est par ailleurs assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

titre du CGI. S'ils sont vendus dans un délai de cinq ans à l'issue de la rénovation lourde s'applique alors la fiscalité précédemment décrite des immeubles neufs, à savoir droits d'enregistrement très réduits et la TVA. En conséquence, la collectivité locale où est situé ledit immeuble ne bénéficie d'aucune recette fiscale, alors même qu'elle a pu faire face à des dépenses pour

Le Gouvernement émet un avis défavorable, puisque cet amendement a pour objet, lors d'une vente d'immeuble neuf, d'affecter aux communes une quote-part du produit net de la TVA correspondant au montant qu'elles auraient perçu

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. » Notre amendement vise à descendre le seuil de publicité à 100 000 euros d'aide fiscale. ne s'agit pas pour nous de donner un volume supplémentaire à tout document retraçant l'aide publique de caractère fiscal. Nous souhaitons cet abaissement tout simplement parce que, de manière unitaire, certains dispositifs ne portent pas sur des versements ou aides très importants.

Nous avons souvent parlé de transparence avec les échanges automatiques d'informations. Cet amendement vise à exclure de la clause de sauvegarde les pays qui n'ont pas conclu d'accord bilatéral ou multilatéral permettant l'échange automatique d'informations avec la France, et ce conformément au standard de l'OCDE.

ne poursuit pas le même objectif que celui qui est prévu à l'article 123 du même code. Le premier concerne la déclaration des comptes bancaires par les institutions financières ; le second cible les situations anti-abus visant les personnes physiques qui délocalisent leurs avoirs afin d'éluder l'impôt. Il s'ensuit que la circonstance qu'il existe un tel accord avec la France est indifférente au regard de l'objectif affiché de la disposition, qui est de s'assurer que la France aura les moyens d'asseoir et de recouvrer l'impôt relatif aux sommes visées à l'article 123 . La parole est à M. le

Je regarde à nouveau le commentaire d'article qui figure dans le rapport de la commission. Nous avons considéré que le champ des exceptions était en pratique extrêmement restreint. La crainte de la commission est que l'article 123 ne devienne à l'avenir quasiment impossible Je vous donne deux exemples. Sur les dix pays concernés par la rectification opérée par l'administration fiscale en 2015, aucun ne figurait sur la liste des États et territoires non coopératifs. Je vous rappelle que le Panama

l'exigence formelle d'un tel accord, suffisante pour activer la clause de sauvegarde du présent article, ne garantit nullement une mise en oeuvre concrète de ce recouvrement. Cet amendement a pour objet d'ajouter un troisième critère, qui permettrait de bénéficier de la clause de sauvegarde du présent article : l'exigence d'avoir conclu un accord bilatéral ou multilatéral avec la France permettant l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale. Je mets aux voix

En vue d'accompagner la volonté de faire des Français des investisseurs en capital, le présent amendement vise à surmonter le paradoxe du PEA-PME, lequel, après un succès populaire, avec plus de 80 000 plans ouverts, a connu un certain reflux, ce nombre étant tombé à 57 700 en décembre 2016. Or, si seulement 5 000 PEA-PME étaient pleinement investis, le montant global de la collecte serait multiplié par deux. L'objet du présent amendement est d'exonérer d'impôt sur les plus-values pour une durée déterminée, à savoir l'année 2018, les cessions de titres ou de parts de FCP ou de SICAV, dès lors que les produits de cessions ainsi réalisées, dans la limite d'un plafond de 75 000 euros, seraient intégralement réinvestis dans un PEA-PME. Cette mesure participera activement au choc d'investissement vers les PME-ETI, dans la ligne de la logique fiscale du Gouvernement. Par ailleurs, elle ne favorisera pas l'optimisation fiscale dans une vision court-termiste, mais, au contraire, servira le financement dynamique des PME. On vise ici le risque plutôt que l'épargne dormante et la rente. La perte de recettes fiscales pour l'État que cet amendement pourrait engendrer est loin d'être avérée, puisque, hors du cadre proposé, aucune plus-value ne sera réalisée. Cette perspective se trouve par ailleurs totalement contredite par la rentrée immédiate de CSG-CRDS dans les caisses de l'État. Cet amendement pose deux difficultés à mon sens. La première, c'est qu'il est rédigé de manière très large. Il va d'ailleurs au-delà de ce que suggère l'objet, qui évoque les cessions de

en recentrant le dispositif incitatif en matière de report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Ce recentrage est proposé en direct et les FCPR ou sociétés de capital-risque sur les sociétés non cotées suivantes : les petites et moyennes entreprises au sens de la définition européenne et les entreprises de taille intermédiaire. Ces entreprises, en effet, ne bénéficient pas du même accès au financement, notamment les marchés, que les grandes entreprises. En vue de leur permettre de poursuivre leur développement, il convient donc d'encourager le financement en fonds propres directement et indirectement les FCPR ou sociétés de capital-risque.

général : en effet, le mécanisme du report d'imposition prévu par l'article 150-0-B du code général des impôts est un dispositif anti-abus visant à mettre fin à des schémas d'optimisation grâce auxquels les cotisants cherchent à échapper à l'imposition des plus-values de cession de cession de valeurs mobilières. Il n'apparaît pas judicieux de vouloir faire de ce dispositif un mécanisme de soutien à l'investissement au capital des PME non cotées. Cela vaut également pour la proposition qui consiste à autoriser le report d'imposition en cas de remploi dans une société non cotée un FCPE ou une SCR. Je ne nie pas l'intérêt des fonds d'investissement, c'est une évidence, mais, pour l'investisseur, il s'agit aussi d'un outil de gestion d'un portefeuille de participations, à distinguer de l'investissement productif. Or si le maintien du report est réservé en cas de remploi dans une société opérationnelle, c'est bien pour ne pas freiner le cycle des investissements productifs normaux. Ce que vous proposez va au-delà, en permettant une entorse à la logique même du dispositif et en autorisant le maintien du report d'imposition en cas de remploi dans de simples sociétés d'investissement, pas nécessairement opérationnelles. Par ailleurs, et d'un point de vue plus général, il ne nous semble pas opportun de mettre en place un régime dérogatoire pour les investisseurs qui choisissent de souscrire des parts de fonds de capital-risque ou d'actions de SCR, dont il ne vous a pas échappé que le régime fiscal est déjà particulièrement favorable. Pour ces raisons, l'avis est défavorable, à moins que vous n'acceptiez, madame la sénatrice, de retirer l'amendement.

Paradoxalement, cela pourrait nuire à la réalisation de travaux si des ventes sont envisagées. Comme l'objectif du dispositif est la réalisation de travaux forestiers, l'obligation de conservation n'a pas de sens dès lors que les travaux sont effectués.

En effet, les frais liés aux ventes de parcelles forestières peuvent représenter 30 % à 50 % de la valeur des biens concernés, ce qui freine, de fait, la restructuration foncière des petits patrimoines.

L'Assemblée nationale, en première lecture du projet de loi de finances pour 2018, a prolongé d'un an, jusqu'au 31 décembre 2018, ce dispositif qui devait expirer au 31 décembre 2017. Le dispositif fiscal Censi-Bouvard soutient la construction de résidences-services destinées aux étudiants ou aux seniors autonomes. Il permet de construire 5 000 habitations principales chaque année. Les contribuables qui en bénéficient, souvent des primo-investisseurs dans le logement, sont issus de la France des classes moyennes. Il représente une alternative équitable au régime fiscal de droit commun de la location meublée professionnelle et non professionnelle, régime qui favorise les contribuables aux taux marginaux d'imposition les plus élevés.

Les classes moyennes ont des difficultés à assurer le premier apport. Au travers de cet amendement, nous proposons

court ! Je n'ai pas entendu d'objection sur le fond, c'est-à-dire sur la situation réelle de l'accession à la propriété des classes moyennes.

Monsieur Janssens, l'amendement n° 167 rectifié

Il est en effet généralement admis que ce sont des difficultés foncières qui engendrent les obstacles à toute construction ambitieuse ou réalisation à grande échelle de logements locatifs sociaux. Pour couler du béton sans caractère social, les choses sont souvent beaucoup plus simples ! Il suffit de regarder l'état de la construction et les données conjoncturelles fournies par l'INSEE

il y a fort à parier que la politique du logement fera partie des éléments de jugement des électeurs le moment venu, aux alentours du printemps 2022. Cela nous amène à préconiser, comme d'autres, une utilisation rationnelle et intelligente des capacités foncières existantes. Aussi, distinguer foncier et bâti dans la réalisation de certaines opérations est une voie qu'il nous convient d'explorer plus avant que cela n'est possible aujourd'hui. Nous pensons même qu'il nous faudrait réfléchir à des dispositifs par lesquels, sous couvert du règlement d'une redevance d'usage, tel terrain appartenant à l'État ou à une personne morale de droit public pourrait être mis en location sous condition d'emploi à la réalisation de logements locatifs sociaux. En tout cas, face à la crise du logement, l'ingénierie sociale et économique nous semble devoir être particulièrement mobilisée, parce que tout n'a manifestement pas été essayé ! Tel est le sens de ces deux amendements et de ce

L'objet de ces sociétés ne peut excéder les compétences des organismes d'HLM qui les ont constituées, ce qui signifie qu'elles ne peuvent réaliser que des opérations de logements sociaux. Nous proposons également que cette exonération s'applique aux cessions réalisées au profit

du champ du prélèvement fiscal unique aux cessions et aux plus-values immobilières ou même mobilières. Cela ne nous est pas paru opportun à ce stade, mais cela ne signifie pas que nous ne regardons pas avec attention ce qui est fait. En matière d'exonérations,

à Mme Christine Lavarde. Cet amendement vise à mettre le dispositif de l'article 16 en cohérence avec les choix opérés par ailleurs en matière d'incitations fiscales à la construction, à savoir, notamment, le dispositif Pinel et le

Face à une demande soutenue, il est nécessaire de créer les conditions d'un choc d'offre, ce qui nécessite, outre des simplifications réglementaires et une lutte accrue contre les recours abusifs, la libération de davantage de foncier. Le dispositif d'abattement exceptionnel sur les plus-values de cessions immobilières introduit par l'article 16 poursuit cet objectif, mais sur un zonage plus restrictif, puisqu'il ne vise que les zones A et A.

pris par le Président de la République d'apporter une réponse différenciée. Par ailleurs, compte tenu du coût substantiel pour les finances publiques de cet abattement applicable aux cessions immobilières, le centrage sur les seules zones les plus tendues A et A paraît indispensable. Madame Lavarde, l'amendement n°

La condition de densification sera considérée comme remplie dès lors que le bâtiment destiné à l'habitation aura un gabarit au moins égal à 80 % du gabarit maximal autorisé, tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. D'autre part, la référence aux constructions de « bâtiments d'habitation collectifs » de préférence aux « locaux destinés à l'habitation » permet de mieux circonscrire la nature des programmes immobiliers visés par la mesure.